madame la présidente.

du Gouvernement ? L'exclusion totale du soja ne nous paraît pas justifiée au regard du risque environnemental qu'il présente par rapport aux autres matières premières en concurrence alimentaire. Un plafonnement semble plus

on a besoin de toutes les productions, dans les limites du raisonnable, en privilégiant bien sûr les productions françaises.

Un taux de 0,70 % dès 2021 représente une position intermédiaire et réaliste en vue d'atteindre le taux de 0,35 % en 2022. Les producteurs partagent ces objectifs. Une entrée en vigueur au 1 janvier 2021 vise à préserver l'effet utile de la mesure : la lutte contre la déforestation importée. En effet, une application au 1 juillet permettrait une utilisation très forte de biocarburants à base de soja,

au renforcement des règles de plafonnement de l'avantage fiscal du soja dès 2021. Cela s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée. Nous avons déposé un sous-amendement rédactionnel et faire en sorte que l'application des règles de plafonnement aux produits pour lesquels la taxe devient éligible le soit dès le 1 janvier 2021.

prévoir une entrée en vigueur de la réduction de 0,7 % dès le 1 janvier 2021 créerait des perturbations dans le bon fonctionnement des filières.

: La parole est à M. Bernard Buis. Cet amendement a pour objet de cibler l'avantage fiscal accordé pour la fourniture d'électricité d'origine renouvelable pour l'alimentation des véhicules électriques sur les exploitants d'infrastructures de recharge ouvertes au public.

n'y ont pas un intérêt direct. Afin d'assurer la mise en oeuvre de cette nouvelle modalité, cet amendement tend à prévoir qu'un décret viendra préciser les obligations de décompte et de transmission d'informations à l'administration, qui permettront d'assurer le respect des conditions de l'avantage fiscal par les exploitants. Quel est l'avis de la commission ? Sur cet amendement,

qui formeront ainsi une troisième filière, aux côtés des essences et des gazoles, et pour lesquels il est fixé un taux cible de 1 %. L'objet de cet amendement est de permettre la comptabilisation des biocarburants issus des filières agricoles françaises dans ce nouvel objectif d'incorporation. Cela répond à un double impératif. D'une part, sans ces biocarburants issus des filières agricoles françaises, la filière « carburéacteurs » sera une filière d'importation, la France ne produisant pas encore suffisamment de biocarburants avancés à destination du secteur de l'aviation. D'autre part, l'exclusion de ces biocarburants est incohérente avec la stratégie nationale sur les protéines végétales issues notamment de colza et de tournesol et le plan Protéines de France Relance. Quel l'avis de la commission ?

ou biocarburants de première génération, puisque l'on parle là des biocarburants de première génération dans le secteur aérien, se ferait au détriment des biocarburants avancés. Il nous semble par ailleurs que cette prise en compte n'ouvrirait probablement aucun débouché nouveau pour ces biocarburants, dans la mesure où la part d'utilisation de ceux-ci dans

M. Pierre Cuypers. Il s'agit d'introduire un tarif réduit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques pour les biocarburants incorporés au fioul domestique. Au contraire des transports routiers et aéronautiques, le recours aux biocarburants pour le chauffage est peu valorisé par les pouvoirs publics. Or la Convention citoyenne pour le climat a adopté le principe de l'interdiction des nouvelles chaudières à fioul à compter du 1 janvier 2022.

vise à permettre le développement de solutions durables à même d'assurer les besoins en chauffage, tout particulièrement dans les zones rurales. Rappelons que le Gouvernement a décidé l'interdiction de chaudières à fioul 100 % fossile à partir du 1 janvier 2022. cet amendement offre donc une solution de substitution sérieuse et cohérente avec les enjeux de transition énergétique. En effet, le fioul domestique est aujourd'hui la troisième énergie de chauffage en France ; il est utilisé par plus de 3,5 millions de ménages vivant essentiellement en maison individuelle, dans des territoires ruraux bien souvent non desservis par des réseaux de chaleur ou de gaz. Cet amendement a donc pour objet la mise en place d'une fiscalité adaptée et incitative pour le déploiement d'un nouveau combustible végétal remplaçant le fioul domestique 100 % fossile.

n° I-154 rectifié. Cet amendement vise à adopter une fiscalité adaptée et incitative pour le déploiement d'un nouveau combustible consistant à remplacer le fioul domestique 100 % fossile par un biofioul contenant jusqu'à 30 % d'ester méthylique d'acide gras, dit « F30 ». Il s'agit de créer pour le F30 une nouvelle ligne fiscale à l'article 265 du code des douanes et de lui appliquer le taux minimal communautaire de TICPE. Le développement de bioliquide renouvelable, par substitution au fioul fossile, contribue à rattraper le retard de la France en matière d'énergie renouvelable. Il peut constituer une évolution provisoire, en attendant de passer à l'étape suivante de 50 % d'introduction d'énergie renouvelable. Enfin, le biofioul répond aux besoins en chauffage des zones rurales. Le fioul domestique est aujourd'hui la troisième énergie de chauffage en France, utilisée par plus de 3,5 millions de ménages, vivant essentiellement dans des maisons individuelles qui ne bénéficient pas d'approvisionnement en gaz de réseau. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas,

cet amendement se rattache au sujet plus large de la rénovation énergétique des bâtiments, priorité clairement définie par le Gouvernement dans le cadre de son plan de relance. Il s'agit en l'occurrence de mettre en place une fiscalité propre pour le déploiement d'un nouveau combustible, remplaçant le fioul domestique 100 % fossile, dont les émissions d'équivalent CO2 sont en deçà de la limite de 250 grammes d'équivalent CO2 par kilowattheure PCI. Il s'agit d'un biofioul contenant jusqu'à 30 % d'ester méthylique d'acide gras, dit « F30 L'objectif de transition écologique imposera par ailleurs une très basse teneur en soufre de ce biofioul, conformément aux objectifs du décret n° 2017-949 du 10 mai 2017. amendement vise à créer une nouvelle ligne fiscale à l'article 265 du code des douanes pour le F30 et à lui appliquer un taux de taxation ne portant pas sur la part renouvelable. En outre, il s'agit de prévoir que la biomasse liquide utilisée en chauffage, l'ester méthylique de colza, ne supporte pas la TICPE, à l'instar de la biomasse solide. Considérant que les chaudières neuves, dites de très haute performance énergique, économisent plus de 30 % de combustible pour un besoin de chauffage équivalent, le consommateur n'en serait globalement pas affecté. De plus, la mesure prévue prend en considération le fait que les travaux de normalisation du F30, actuellement engagés sous l'égide de la direction générale de l'énergie par le Bureau de normalisation du pétrole sous mandat Afnor, sont amenés à aboutir après la publication de ce L'objectif principal de cet amendement est de permettre une alternative, plus particulièrement en zone rurale- c'est l'un de ses points forts -, en cohérence avec la décision du Gouvernement d'interdire l'installation de chaudières à fioul 100 % fossile à partir du 1 janvier 2022. À cette fin, il convient de soutenir activement la mise en place d'un processus rapide de remplacement du fioul domestique fossile par un bioliquide renouvelable permettant de répondre à ces nouveaux critères d'émissions de gaz à effet de serre. La perte fiscale est très relative, puisque seules les nouvelles chaudières installées à partir de 2022 seront tenues à l'utilisation de ce biofioul, soit environ 35 000 chaudières par an, ce qui représente une consommation en année pleine de 26 000 mètres cubes et un impact fiscal de 1,3 million d'euros en 2022. en 2022. Le développement de bioliquide renouvelable est encouragé par la directive UE 2018/2001, et l'essor d'un bioliquide en France par substitution du fioul fossile contribuera à rattraper le retard français en matière d'énergie renouvelable.

est l'avis de la commission ? À ma connaissance, le biofioul n'est pas pour le moment commercialisé en France

dans cet hémicycle, je rappelle que le droit de l'Union européenne encadre strictement le recours au tarif réduit de TICPE. D'une part, la réduction doit s'appliquer à raison de la part réelle d'énergies renouvelables ou à une part minimale contenue dans le produit.

que le développement de moyens de chauffage alternatifs au fioul fait partie des priorités environnementales du Gouvernement. Même si elle peut parfois être moins polluante, il s'agit néanmoins d'une d'une énergie coûteuse, qui est soumise par ailleurs aux aléas du prix du baril. Par ailleurs, le Gouvernement a mis en place une prime à la conversion des chaudières au fioul avec un objectif simple et ambitieux remplacer en deux ans 600 000 chaudières par des équipements à haute performance environnementale. Cette prime cumulative avec les autres dispositifs permettra d'assurer la conversion du parc et de diminuer la facture des ménages. Pour des raisons d'inconventionnalité et parce que cela ne lui

Il s'agit d'inciter la CRE à supprimer la majoration de la composante de soutirage du Turpe spécifique sur la part autoproduite, afin d'alléger de manière d'autant plus significative les charges sur les projets d'autoconsommation collective. Le coût supplémentaire dans le budget pour 2021 serait de l'ordre de 84 000 euros. Je le rappelle, les projets d'autoconsommation collective ne représentent en 2020 que 0,003 % de la puissance installée d'énergies renouvelables en France. Pourtant, seulement 17,8 % de la consommation finale brute d'énergie provenait d'EnR en 2019, le développement de ces projets est essentiel si la France veut atteindre son objectif de 33 % de la consommation finale brute d'énergie provenant d'EnR d'ici à 2030. objectifs. D'abord, il vise à encourager la création de projets d'autoconsommation collective en établissant un cadre réglementaire plus favorable sans devoir supporter de charges disproportionnées, conformément à la directive Si les projets d'autoconsommation individuelle sont rentables grâce à des avantages fiscaux, ce n'est pour l'instant pas le cas des projets d'autoconsommation collective. Ensuite, il tend à améliorer l'acceptation sociale des projets d'énergie renouvelable en favorisant la coconstruction entre citoyens et acteurs d'un même territoire : entreprises, bailleurs sociaux, collectivités le rappelle, 70 % des projets privés d'éoliennes sont freinés par des recours au tribunal par les locaux. Enfin, il vise à augmenter les rendements des projets d'EnR à l'échelle locale. Pour 1 euro investi, 2,5 euros profitent directement au territoire. De tels projets pourraient donc être un catalyseur essentiel de la transition énergétique des territoires.

en établissant un cadre réglementaire beaucoup plus favorable qu'actuellement. L'amendement vise à exonérer de taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité la part d'électricité autoproduite par les projets d'autoconsommation collective au même titre que

L'absence de renouvellement des concessions hydroélectriques, au nombre d'une vingtaine à ce jour, aboutissait à un manque à gagner pour les finances publiques du fait de l'absence de versement de la redevance proportionnelle. Pour y remédier, la loi de finances pour 2019 a instauré une disposition visant à créer une redevance, au bénéfice de l'État et des collectivités locales, pour ces concessions hydroélectriques exploitées sous le régime des « délais glissants

de calcul retenu, sur un rendement manifestement très inférieur aux estimations effectuées et ne permet pas un contrôle effectif de la part des collectivités bénéficiaires.

Or la plus importante de France, Bissorte/Super-Bissorte, n'a donné lieu qu'à une notification de 162 000 euros, certaines ne donnant lieu à aucun versement. Cela résulte du contenu du décret du 28 juillet 2019, qui n'est pas totalement fidèle à la loi votée par la représentation nationale. Toujours dans cette note, la Cour des comptes relève qu'il existe donc certainement « une marge pour réviser à la hausse le niveau des redevances proportionnelles aux recettes applicable aux concessions en délai glissant Elle invite le Gouvernement à procéder à l'examen de cette situation : « Si une telle marge était confirmée, il conviendrait d'envisager de réviser la formule de calcul de la redevance, afin de valoriser aux mieux le patrimoine de l'État. » Au regard de ces observations et du constat qu'il n'existe pas de méthode indiscutable permettant d'évaluer la rentabilité d'une concession, nous proposons d'ores et déjà de supprimer la référence au critère des bénéfices pour le calcul de la nouvelle redevance. Une assiette de la redevance basée sur les recettes de la concession permet d'aboutir à un système plus adapté à la situation de chaque concession et d'assurer un rendement correct au bénéfice de l'État et des collectivités locales. L'amendement vise par ailleurs à instaurer un droit de communication aux collectivités territoriales concernées sur les données financières des concessions.

Enfin, les informations sur les résultats financiers d'une concession relèvent du secret fiscal, ainsi que du secret industriel et commercial. Elles ne peuvent donc pas être communiquées aux collectivités et groupements bénéficiaires, comme le proposent les auteurs de l'amendement. L'adoption de cet amendement risquerait de fragiliser les concessions hydroélectriques.

en particulier celles qui assurent le trafic transmanche, qui sont confrontées au problème du Brexit. La situation, notamment de la compagnie Brittany Ferries, est particulièrement critique.

L'enjeu est réel. Il s'agit de prolonger une mesure de soutien à la filière de biogazole, durement frappée par la chute de 75 % de la consommation de gazole au printemps dernier. Un tel dispositif ne coûte rien.

Dans le contexte du précédent confinement lié à la covid-19, la troisième loi de finances rectificative pour 2020 comportait, dans le cas de la taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants, une mesure de majoration de 20 % de la comptabilisation des esters méthyliques d'acides gras présentant une bonne résistance au froid. L'objectif était de permettre l'écoulement de biocarburants dits « de qualité hiver » demeurés invendus pendant la période de confinement. En effet, la filière avait maintenu sa production pour continuer à cogénérer de la protéine végétale et préserver ainsi la chaîne alimentaire. Alors que ce dispositif de taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants devait avoir un plein effet durant cette fin d'année, de septembre à décembre, le nouveau confinement intervenu en octobre vient changer la donne. Dans ce contexte, cet amendement vise à prolonger la mesure jusqu'à la fin du premier trimestre de 2021.

les SDIS de cette taxe permettrait d'orienter davantage leurs dépenses vers l'investissement et, donc, de favoriser l'efficacité de leurs interventions.

par exemple les sections ou associations de la Croix-Rouge française ou de la Fédération française de sauvetage et de secourisme. Ces organismes reposent largement sur le bénévolat et sont confrontés à un manque de moyens pour répondre aux nombreuses sollicitations dont ils font l'objet de la part des pouvoirs publics, des collectivités locales ou des organisateurs d'événements. Au-delà de leurs ressources propres, ces associations bénéficient de subventions publiques, mais l'évolution de ces dernières ne permet pas de répondre aux besoins croissants. Nous proposons donc, par cet amendement, de mieux les soutenir dans l'exercice de leurs missions en les exonérant de TICPE.

utilisée pour les interventions des véhicules des sapeurs-pompiers. Ce remboursement existe déjà pour les services de transports publics routiers en commun de voyageurs. Les sapeurs-pompiers concourant à l'exécution d'un service public vital, il semble cohérent qu'ils puissent également en bénéficier, afin de favoriser leurs dépenses d'investissement grâce au redéploiement de ces crédits.

Il s'agit en effet d'une niche fiscale nuisible au climat, mais aussi génératrice d'externalités négatives fortes pour les riverains des ports, avec des incidences sur la santé publique et l'environnement. D'après une étude menée par l'ONG Transport & Environnement, l'ensemble des navires de croisière qui font escale à Marseille émettent autant d'oxyde d'azote que le quart des voitures qui composent la flotte automobile de la ville.

Enfin, concernant les particules fines, dans des quartiers résidentiels de la ville aux abords du port, l'air est jusqu'à vingt fois plus pollué. Chaque année, en Europe, ces émissions du transport maritime causent près de 60 000 morts et coûtent 58 milliards d'euros aux services de santé. Il est donc temps d'en finir avec cette niche fiscale nocive qui bénéficie au secteur des croisières, d'immenses paquebots, alors que son impact négatif sur la santé et l'environnement n'est plus à démontrer.

La fiscalité des produits énergétiques est harmonisée par le droit européen, qui ne permet des exonérations que pour les usages commerciaux et industriels ou pour les besoins des autorités publiques.

au sein de l'Union européenne. Il est difficile de vouloir à la fois éviter que certains pays, de manière totalement unilatérale, pratiquent une fiscalité basse dans des domaines d'intérêt général

pour contraindre les États à rester dans un corridor de fiscalité et éviter des comportements regrettables au sein de l'Union européenne.

que des pratiques qui ont un impact énorme sur le climat, la santé et la biodiversité bénéficient de fortes niches fiscales alors qu'un tout petit geste est

En revanche, soucieux de favoriser durablement les solutions de mobilité plus respectueuses de l'environnement, le Gouvernement a soutenu, dans le cadre de l'examen du présent projet de loi de finances à l'Assemblée nationale, la prorogation du dispositif.

est de stabiliser les émissions de carbone au même niveau à partir de 2020. Le présent amendement respecte cet engagement du Gouvernement.

carbone. Rappelons que l'article 56 de la loi de finances pour 2019 avait instauré un dispositif de même nature pour le transport maritime.

dans l'objectif de renouveler et de moderniser la flotte. Cette exonération, soumise à une condition de réinvestissement de la plus-value dans un bateau plus récent ou plus capacitaire, est aujourd'hui plafonnée à 100 000 euros par cession. Cette limitation constitue une exception par rapport aux autres pays européens concernés par le transport fluvial, notamment les Pays-Bas, la Belgique et l'Allemagne, dont le régime d'exonération ne prévoit pas de plafond. Cet amendement vise donc à supprimer le plafond afin de favoriser le renouvellement de la flotte et d'améliorer la compétitivité du transport fluvial face à la concurrence européenne. Il tend également à améliorer sa compétitivité face à la route, dans une logique de report modal vers la voie d'eau, bien moins polluante et plus capacitaire,

Il nous paraît également suffisamment incitatif et favorable au développement du transport fluvial de marchandises. Supprimer le plafond de cession conduirait en pratique à exclure les cessions les plus importantes de l'encadrement européen, qui assure sa compatibilité avec la réglementation des aides d'État.

concernant cet argument de justice, vous n'avez pas non plus réagi sur le fait que le secteur de l'aviation d'affaires, des jets privés, a été oublié en 2020.

qui échappent à cette contribution au climat. Comment voulez-vous faire entendre à une personne qui prend son véhicule diesel tous les jours qu'elle va payer une taxe supplémentaire sur son gazole si ceux qui jouissent de grands avantages n'en paient pas ? C'est impossible

l'avis du Gouvernement ?

représente des milliards d'euros perdus, au détriment des particuliers et des collectivités territoriales, avec des conséquences majeures aux niveaux environnemental, social et sanitaire. Cet abandon coûteux a fait perdre à l'Afitf une ressource pérenne de 1 milliard d'euros annuels. La compensation de cette perte de ressources n'a été que partielle, avec l'affectation d'une partie de la TICPE au budget de l'Afitf, à hauteur de 400 millions d'euros Moduler la taxe d'aménagement du territoire pour instaurer une contribution du transport routier de marchandises permettra de faire contribuer l'ensemble des poids lourds, y compris les pavillons étrangers, à l'amélioration des infrastructures de transport, en accroissant les moyens de l'Afitf. de l'Afitf. Nous proposons, pour les poids lourds, autocars et véhicules assimilés de plus de 7,5 tonnes, un montant de taxe augmenté de 50 % par rapport à la taxe perçue par les autres véhicules.

ne pas proroger les contrats actuels et de tenter de les renégocier, en appelant à une grande concertation, que Vincent Delahaye a nommée « Défense des autoroutes ». L'augmentation de la taxe d'aménagement du territoire permettrait d'engager cette discussion.

schémas anciens. Nous proposons d'augmenter la taxe d'aménagement du territoire due par les concessionnaires d'autoroutes à raison du nombre de kilomètres parcourus par les usagers.

tonnes, avec un coefficient multiplicateur de trois par rapport à la taxe perçue pour les autres véhicules. Une telle mesure permettra de faire contribuer l'ensemble des poids lourds, y compris les pavillons étrangers, à l'amélioration des infrastructures de transport en accroissant les moyens de l'Afitf, rapprochant ainsi du scénario 3 du Conseil d'orientation des infrastructures.

Voilà une manière simple et efficace de renflouer les caisses de l'Afitf et de pénaliser un mode de transport particulièrement polluant

estime qu'une indexation sur l'inflation n'est pas de nature à modifier l'équilibre des contrats, dès lors que l'augmentation annuelle des tarifs est supérieure à l'inflation et que ceux-ci augmentent, de toute façon, plus vite que la taxe d'aménagement du territoire. Au regard de ces éléments, rien ne justifie que la taxe due ne soit majorée qu'à hauteur de 70 % de l'inflation. Le présent amendement de Vincent Delahaye vise à indexer le tarif de la taxe d'aménagement du territoire sur l'inflation, ni plus ni moins. Quel

au Gouvernement de solliciter l'avis du Conseil d'État sur la légalité de ces contrats- je dis bien la « légalité » de ces contrats -au vu de l'équilibre économique

rectifié. Nous proposons un lissage sur trois ans de la hausse du tarif de la TICPE applicable à l'essence d'aviation utilisée pour l'aviation légère et sportive. Actuellement à l'arrêt complet du fait de la crise sanitaire et des restrictions de déplacement, l'aviation légère et sportive ne pourra supporter une hausse d'une telle ampleur d'un seul coup. vise également à affecter ce surplus de TICPE à la transformation énergétique de l'aviation légère et sportive. Ces activités aériennes font office de précurseur dans la transition énergétique du secteur aéronautique. L'aviation légère et sportive joue aussi un rôle déterminant dans la formation des acteurs du secteur de l'aérien. Il n'est donc pas souhaitable de la fragiliser encore plus avec une hausse aussi brutale de la TICPE. La parole

Elle a aussi un rôle dans la formation des acteurs du secteur de l'aérien. Pourraient être envisagés notamment une subvention de transition écologique vers l'avion à moteur électrique pour la formation au pilotage au pilotage de début, un bonus écologique pour les avions légers remotorisés avec un moteur thermique de nouvelle génération à faibles émissions de CO2 une prime à la conversion pour remplacer les aéronefs légers anciens par des aéronefs de nouvelle génération.

pour l'essence d'aviation sur deux ans est cohérente avec la proposition de la Convention citoyenne pour le climat. Il nous semble qu'une augmentation de la taxe sur trois ans nuirait à l'objectif de réduction des émissions de dioxyde de carbone à court terme, sur lequel le Gouvernement s'est engagé.

est à M. André Guiol. Face à la crise sanitaire et désormais économique, l'augmentation de la TICPE prévue pour le GNR pénaliserait de nombreuses entreprises dans les secteurs agricole,

Je vous remercie

Pour faire face aux difficultés rencontrées par les opérateurs, des mesures favorables aux entreprises ont été adoptées, notamment pour celles du secteur du bâtiment et des travaux publics, ainsi que pour d'autres utilisateurs de gazole non routier. Il ne nous semble pas souhaitable de revenir sur cet équilibre, qui a fait l'objet d'une concertation avec les professionnels et qui garantit l'acceptabilité de la suppression de la dépense fiscale liée au GNR.

dans la mesure où ce secteur n'a pas été soumis aux évolutions du tarif du gazole issu de la trajectoire carbone. Par ailleurs, afin d'améliorer la trésorerie des entreprises de transport dans le cadre de la crise sanitaire, je rappelle que la périodicité du remboursement partiel est devenue trimestrielle, alors qu'elle était semestrielle. Aussi, les transporteurs n'acquitteront pas de taxe à l'essieu en 2021.

La loi de finances rectificative de juillet 2020 a mis en place deux dispositifs destinés à entrer en vigueur le 1juillet 2021 : d'abord, un registre de suivi, afin de s'assurer que le carburant employé

Les travaux d'élaboration de cette liste n'ont toujours pas abouti à ce jour en raison de l'incongruité de cet objet : un matériel en tant que tel ne peut présumer, par ses seules caractéristiques, de l'usage qui en sera fait. C'est la raison pour laquelle, conformément à l'article 8

en l'état de la loi, pour l'exercice d'activités de travaux publics, seules les entreprises agricoles devront tenir le registre de suivi de ces travaux et s'assurer que le donneur d'ordre le tient aussi, sous peine d'une amende de 10 000 euros en cas d'absence de registre ou d'une amende de 300 à 3 000 euros en cas d'inexactitudes sur ce registre. Cette différence de traitement entre une entreprise agricole et une entreprise de travaux publics porte indubitablement atteinte à une concurrence saine et loyale entre opérateurs, puisqu'elle fait peser des obligations et contraintes uniquement sur les entreprises agricoles du seul fait de la nature de leur activité principale. Tels sont les motifs qui justifient cet amendement. Quel est l'avis de la commission ?

était adopté, nous exposerait à des demandes reconventionnelles, qui auraient pour effet d'affaiblir à terme la stratégie environnementale du Gouvernement en matière de soutien aux fabricants de matériel propre. Je rappelle par ailleurs que les entreprises produisant des substances minérales solides peuvent bénéficier de la déduction à raison des engins utilisant des carburants respectueux de l'environnement.

Ledit article a mis en place un registre de suivi des travaux non agricoles et non forestiers, afin d'améliorer le contrôle des volumes de gazole non routier éligibles au remboursement partiel de TICPE.

leur code NAF ou leur forme sociale, devraient être éligibles au remboursement partiel de TICPE, dès lors qu'elles utilisent du GNR pour réaliser des travaux agricoles ou forestiers. À titre d'illustration, le carburant utilisé dans un tracteur agricole pour le transport de matières agricoles en dehors de l'activité de récolte n'est pas éligible à l'emploi de gazole non routier et nécessite donc l'emploi de gazole blanc- on va vraiment dans la complexité. À l'inverse, le carburant utilisé par une minipelle dans le cadre de travaux forestiers peut bénéficier, lui, de l'emploi du GNR et même de gazole agricole. Le concept même de cette liste est contraire aux principes du droit communautaire. Il

injecté dans les réseaux, dont la traçabilité est assurée par les garanties d'origine. Cette mesure serait neutre pour le budget de l'État, l'exonération ciblée se substituant à la baisse générale du taux de la taxe. Il est logique que le gaz renouvelable soit exonéré de TICGN, puisque, depuis 2014, cette taxe est par construction constituée d'une composante carbone, la contribution climat-énergie, qui vise à créer un différentiel de prix entre les énergies fossiles et les énergies renouvelables pour favoriser le développement de ces dernières. Le biométhane apporte en outre de nombreux bénéfices environnementaux, sociaux et économiques, qui sont

La loi de finances pour 2020 a rationalisé et simplifié le régime fiscal du gaz. Son article 67 prévoit en effet de forfaitiser l'exonération de la TICGN en appliquant une baisse de la taxe en fonction de la part de biogaz injecté dans les réseaux pour l'ensemble des consommateurs de gaz, qu'ils aient souscrit une offre verte ou non. L'application de telles dispositions ne permettra pas de différencier, sur le plan fiscal, les offres de gaz fossile et les offres de gaz vert, d'ores et déjà moins compétitives du fait de la chute du prix des énergies fossiles. De telles dispositions obéreraient d'autant plus la compétitivité des réseaux de chaleur renouvelable alimentés notamment par du biogaz, alors même que la filière est aujourd'hui en difficulté. Elles iraient par ailleurs à rebours des aspirations actuelles des industriels, collectivités et particuliers souhaitant privilégier les énergies renouvelables par rapport aux énergies fossiles. assurer une taxation différenciée des énergies renouvelables et des énergies fossiles, il apparaît donc pertinent de maintenir une exonération ciblée de la TICGN pour les consommations volontaires de gaz renouvelable injecté dans les réseaux, dont la traçabilité est assurée par les garanties d'origine.

la TICGN pour les consommations volontaires de gaz renouvelable injecté dans les réseaux, dont la traçabilité est assurée par les garanties d'origine.

d'exonération totale du biogaz injecté dans les réseaux. Je n'y suis pas favorable, car, dans un contexte de forte interconnexion des réseaux, l'application de l'exonération

On ne peut que le regretter, car les biocarburants aéronautiques constituent une solution précieuse pour décarboner les avions, la seule solution à court terme en l'absence de propulsion aboutie qui fonctionnerait à l'électricité ou à l'hydrogène. je rappelle que leurs émissions de gaz à effet de serre sont parfois inférieures de 90 % à celles du kérosène classique.

dénonce ainsi un pilotage incohérent, avec, d'un côté, de l'argent consacré à la transition écologique et, de l'autre, des investissements défavorables au climat. Alors que le Conseil d'État appelle le Gouvernement à justifier de ses efforts pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à cet amendement, attendu par le secteur associatif, permettrait enfin de clarifier le message politique, en sortant d'un soutien assumé et permanent aux économies carbonées dans le secteur des transports. l'amendement n° I-934. Cet amendement, que nous déposons chaque année, vise à supprimer l'exonération de taxe intérieure de consommation sur l'ensemble des vols intérieurs. L'exonération fiscale du kérosène est une aberration écologique. Alors que nous sommes invités par la Convention citoyenne pour le climat à réduire nos vols intérieurs quand il existe une alternative ferrée rapide, commençons par supprimer cette exonération absurde en France.

C'est le moment, plus que jamais, de supprimer cette exonération. Ce serait un juste retour pour une entreprise qui ne s'est vu imposer aucune contrepartie écologique ou sociale jusqu'à présent. Si posséder sa propre compagnie aérienne est indispensable pour la souveraineté de la France, alors nationalisons Air France et cessons d'allonger les milliards sans regard

provoquent une pollution massive des eaux, des sols et des eaux souterraines- l'eau que nous buvons, je vous le rappelle. Pour autant, ils sont largement épargnés par des mécanismes financiers qui pourraient inciter à réduire leur utilisation. Il s'agit, ici, de refléter le coût réel des intrants chimiques pour la société. J'ai bien conscience que réduire notre dépendance aux engrais est un sujet délicat, mais c'est un sujet auquel nous devons nous atteler sans tarder, eu égard aux impacts sanitaires et environnementaux Les producteurs d'engrais sont soumis à la taxe générale sur les activités polluantes, la TGAP, du fait des émissions engendrées par ce secteur. Toutefois, leur contribution reste infime, car les seuils d'émissions de polluants à partir desquels les entreprises sont taxées sont beaucoup trop élevés

qui se combinent dans l'atmosphère pour former des particules fines. On observe effectivement des pics de pollution lors des épandages, et 55 % des particules fines sont dues à l'activité agricole. Les composés sont également responsables de l'eutrophisation des milieux aquatiques. Ce sont là des atteintes graves aux écosystèmes.

du modèle agricole vers une gestion plus respectueuse de la santé humaine et de la nature dans sa globalité. Les surplus d'azote constituent un problème écologique majeur. C'est pourquoi cet amendement propose d'inclure, dans la TGAP, les émissions d'ammoniac.

par les associations agréées de surveillance de la qualité de l'air, le réseau Atmo France, concernant l'impact sur la qualité de l'air d'un certain nombre de dispositifs d'épandage d'engrais ou d'utilisation de produits phytosanitaires dans le secteur

explication de vote. Je voudrais rappeler que, en 2016, les secteurs des produits chimiques, des engrais et des matières plastiques ont contribué seulement à hauteur de 6,7 millions d'euros, ce qui ne représente que 0,09 % de leur valeur ajoutée. Un rapport de l'inspection générale des finances de 2018 conclut qu'au taux actuel de taxation la TGAP n'est pas susceptible d'influencer les décisions d'investissement des industriels. Pourtant, les implications de la production d'engrais de synthèse sur la qualité de l'air et la crise climatique justifieraient une approche tournée vers une taxe comportementale.

fortement liées aux engrais azotés de synthèse. Le constat est inquiétant : alors que les pollutions industrielles de l'eau sont en recul, les pollutions agricoles se maintiennent, en particulier avec les nitrates et les pesticides. L'objet L'objet de cet amendement est donc d'inclure l'azote de synthèse dans l'assiette de la redevance pour pollutions diffuses, dont doivent s'acquitter les agriculteurs.

Les engrais azotés de synthèse ont un impact avéré sur la vie des sols, mais aussi sur la qualité de l'eau, alors même que la France peine à appliquer la directive Nitrates. Ce fléau, nous le payons lourdement en Bretagne. L'impact des engrais minéraux sur l'environnement n'étant plus à démontrer, cette taxation permettrait d'influencer les pratiques, en participant au financement de la transition agroécologique. Le présent amendement tend donc à inclure l'azote de synthèse dans l'assiette de la redevance pour pollutions diffuses. Pour éviter un impact négatif de cette taxation sur le revenu des exploitations agricoles, il convient de mettre en place, en parallèle, de très fortes mesures d'accompagnement au changement de pratiques. Je pense notamment au plan Protéines ou au programme de reconquête des haies.

et limiter les besoins en engrais azotés. De même, il faudra renforcer le soutien à la conversion à l'agriculture biologique ou encore aux systèmes herbagers. Les auteurs de cet amendement estiment également que les ressources liées à cette redevance

Il est défendu.

contenant un ou plusieurs micropolluants à compter du 1 juillet 2021. Des produits comme certains médicaments, biocides, même ménagers, produits cosmétiques ou d'hygiène seraient concernés. est identique aux précédents, je vais tout de même développer un argumentaire, car le sujet est important. Par cet amendement, nous souhaitons tendre à la dépollution des milieux aquatiques. La pollution de ces milieux est notamment le fait des micropolluants, des substances issues de produits commerciaux ou industriels, composés organiques ou métalliques. Ils méritent d'autant plus notre attention qu'ils sont susceptibles d'avoir une action toxique pour l'homme et les organismes aquatiques, y compris à des concentrations très faibles dans l'eau. Ces micropolluants sont courants : certains médicaments, biocides ménagers, produits cosmétiques ou d'hygiène en contiennent. L'Agence européenne des produits chimiques en dénombrait plus de 20 000 en mai 2018, dans le cadre du règlement Reach. Plusieurs centaines de nouvelles substances sont mises sur le marché chaque année par les industriels. Notre réponse contre ces micropolluants doit comporter deux volets

contenant un ou plusieurs micropolluants, à compter du 1 juillet 2021. Dans les faits, nous souhaitons appliquer un taux modulé selon la nocivité de la substance indésirable et cumulable selon le nombre de substances. Ce taux reste raisonnable, entre 0,5 % et 1,5 % du prix du produit,

Elle permettrait également de mobiliser de nouveaux financements collectés par les agences de l'eau pour soutenir de nouvelles actions des services publics de gestion de l'eau sur l'ensemble du territoire national. Enfin, pour éviter toute contestation sur la nocivité des substances, nous précisons que les micropolluants concernés figurent dans les listes de vigilance d'ores et déjà existantes aux niveaux français et européen.

une nouvelle redevance, à laquelle les industriels qui importent des médicaments, des biocides, des produits cosmétiques ou des produits d'hygiène contenant un ou plusieurs micropolluants seraient assujettis à partir du 1 juillet 2021. Il est prévu que le taux de cette redevance soit fixé par les agences et offices l'eau pour l'ensemble du territoire national.

Cet amendement vise à supprimer une disposition introduite par la loi de finances pour 2020, qui permet de déplafonner le remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel pour les exploitants agricoles. Cette mesure bénéficie prioritairement au chauffage des serres de maraîchage. Depuis son entrée en vigueur, la production sous serre visant à produire des légumes de contre-saison, en particulier des tomates, à l'aide de chauffage au gaz naturel est donc soutenue financièrement : elle bénéficie désormais d'une aide d'environ 25 000 euros par hectare tous les ans. Auparavant, le remboursement était plafonné à 20 000 euros tous les trois ans. Notre amendement vise à revenir sur cette mesure, qui contrevient à l'objectif d'une fiscalité écologique et d'une transition écologique de l'agriculture. L'argent public,

Cet amendement vise à faciliter la mise en oeuvre de la loi de transition énergétique en faisant en sorte que les collectivités territoriales, en particulier les régions, puissent bénéficier d'une part de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE). Le coût de mise en oeuvre d'un certain nombre de dispositifs est extrêmement lourd

ou d'incitation visant à agir sur les comportements. Son affectation aux actions permettant de respecter nos engagements en faveur du climat et de répondre à l'urgence climatique est une question centrale. En outre, la condition indispensable de son acceptabilité sociale. La fiscalité environnementale doit également bénéficier aux collectivités- c'est l'objet de cet amendement -, car elles ont un grand rôle à jouer dans la transition écologique et dans l'amélioration de la résilience des territoires, par le développement d'une économie locale.

des volets énergie des schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (Sraddet) et des schémas régionaux climat-air-énergie (SRCAE) doivent permettre de structurer une mise en mouvement généralisée des territoires en faveur de la transition énergétique.

Si l'élaboration d'un plan ou d'un schéma coûte environ 1 euro par habitant, sa mise en oeuvre à l'échelle du territoire coûte 100 à 200 euros par habitant.

un transfert supplémentaire de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques grèverait davantage encore cette ressource fiscale, alors même que la consommation de carburant baisse en 2020. Enfin, je rappelle que le plan de relance prévoit de consacrer un effort sans précédent à la transition écologique.

Cet amendement vise à attribuer une partie du produit de la TICPE revenant à l'État aux communautés de communes pour le financement des services de mobilité

Cet amendement est d'autant plus important que la crise sanitaire actuelle, qui induira une baisse importante des recettes fiscales des établissements publics de coopération intercommunale l'année prochaine, pourrait désinciter les communautés de communes à se saisir de cette compétence. C'est pourquoi il convient d'attribuer aux communautés de communes qui, exerçant la compétence d'organisation de la mobilité, ne perçoivent pas de versement mobilité, une fraction de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques pour financer la mise en place

du Gouvernement ? Nous sommes conscients de la nécessité de compenser les effets de la réforme engagée par la loi d'orientation des mobilités. Cependant, les attributions de fractions de TICPE relèvent, à titre principal, du financement des transferts de compétences de l'État aux collectivités territoriales dans le cadre de la fiscalité transférée. Élargir le financement de la politique de mobilité des collectivités territoriales par le biais de la TICPE pourrait fragiliser cette ressource. En outre, une telle mesure nuirait à la lisibilité et à la prévisibilité de cette ressource fiscale, à la fois pour l'État et pour les collectivités.